L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à M. Christian Klinger, auteur de

à l'échelle de la CEA. Le projet de création d'une ligue Alsace était donc en cours et avait obtenu l'accord de l'ancienne équipe dirigeante de la FFT et du ministère chargé des sports.

les circonscriptions administratives de l'État dans les deux départements ne sont pas modifiées. Les services préfectoraux, d'une part, et ceux de l'éducation nationale, d'autre part, demeurent l'échelon départemental. Dans le domaine du sport, monsieur le sénateur, l'article 5 de cette loi prévoit que « les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la collectivité européenne d'Alsace ». Il s'agit donc pour ces organes infrarégionaux de trouver une place dans l'organisation territoriale de la région Grand Est. En l'occurrence, l'annexe du code du sport prévoit déjà la possibilité pour des fédérations sportives agréées de solliciter auprès du ministère chargé des sports une dérogation pour que le ressort territorial des ligues régionales ou des comités départementaux diffère de celui des services déconcentrés du ministère. Il s'agit ainsi de créer un régime d'exception. En outre, le code du sport précise que cette dérogation est envisageable, sous réserve de justification et en l'absence d'opposition motivée du ministère chargé des sports. Mme la ministre chargée des sports le confirme régulièrement, ce cadre réglementaire préexistant dans le code du sport permet à la loi de du 2 août 2019 de trouver sa pleine application sans qu'un nouveau décret d'application soit nécessaire. Dans ce contexte, la Fédération française française de tennis avait initialement envisagé de saisir le ministère chargé des sports d'une demande de création d'une ligue régionale d'Alsace de tennis, et le ministère avait confirmé qu'il examinerait toute demande motivée que la fédération lui adresserait en ce sens, l'organisation territoriale des fédérations relevant de la responsabilité souveraine du mouvement sportif,

Le Pass'Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant, dont l'objectif est de financer l'inscription dans une structure sportive. Il s'adresse aux enfants de 6 à 17 ans, bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. On estime que ce dispositif permet l'inscription sportive de 5,4 millions d'enfants chaque année. Cependant, on note que le Pass'Sport ne peut être utilisé qu'auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive et, dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes les associations sportives agréées participant au dispositif. Or, en milieu rural, des associations ne sont pas affiliées à une fédération sportive. Je pense notamment

de 100 millions d'euros, et ce budget sera reconduit dans le projet de loi de finances pour 2022. Il s'agit là d'une véritable avancée, qui illustre l'engagement du Gouvernement pour démocratiser l'accès au sport et la pratique sportive. Ces 100 millions d'euros servent à soutenir la prise de licence dans les clubs sportifs, à favoriser la reprise des activités

principalement été adressé aux associations affiliées et aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des sports, ce qui représente plus de 150 000 associations sportives. Il a également été ouvert aux associations bénéficiant d'un agrément sport ou jeunesse éducation populaire délivré par le préfet,

que pour l'affiliation aux associations sportives et aux fédérations. Ce dispositif s'applique naturellement sur l'ensemble du territoire national. Les associations sportives, qu'elles se trouvent en milieu rural ou non, ont la possibilité de s'affilier à une ou plusieurs fédérations sportives

entrer sur un terrain, quand bien même l'activité a lieu en plein air. Le décret publié le 7 août dernier prévoit que le contrôle des données est fait une fois et que les données ne sont pas conservées, tant et si bien que les associations doivent contrôler le passe sanitaire à chaque début d'entraînement. Je relève que, dans la presse, un certain nombre de responsables de fédérations ont fait état des difficultés posées par le dispositif, notamment parce qu'il n'appartient pas aux bénévoles de mener ce type d'activité et que ceux-ci ne peuvent pas

Le contrôle du passe sanitaire est confié selon l'organisation la plus pertinente définie à l'échelon local aux personnes chargées de contrôler l'accès à un équipement sportif ou aux bénévoles ou professionnels qui organisent l'activité sportive au sein du club. Dans le domaine sportif, les clubs connaissent bien leurs membres, leur identité

En conséquence, si le passe sanitaire doit être systématiquement contrôlé pour la pratique sportive, le pragmatisme de terrain pour les adhérents possédant un schéma vaccinal complet doit être de mise. En ce qui concerne les jeunes licenciés qui auront 12 ans dans les semaines à venir, le passe sanitaire leur sera applicable à 12 ans et 2 mois

d'État, vous avez rappelé des éléments que l'on connaît déjà ... Vous parlez de pragmatisme, mais j'aurais voulu une réponse claire pour les associations : peuvent-elles, ou non, constituer une liste avec les adhérents qu'elles ont déjà contrôlés ? En l'état, c'est le décret qui s'applique

Ce secteur rassemble un grand nombre d'établissements ; je citerai en particulier le cas de l'institut La Teppe, dans mon département de la Drôme, spécialisé dans le traitement de l'épilepsie. trois impacts négatifs majeurs. Le premier impact est financier. Les décisions issues des accords du Ségur de la santé ont été transposées pour le personnel non médical sans compensation financière suffisante pour les Ces nouvelles dispositions prévoient une revalorisation des salaires à hauteur de 238 euros bruts par mois, qui entraîne un surcoût important en termes de charges sociales patronales, ce qui met en difficulté financière ces établissements. impact touche l'attractivité des maisons de santé, en particulier pour les personnels médicaux. Ces derniers ayant connaissance d'une revalorisation des salaires dans le secteur public demandent leur transfert dans des établissements de ce secteur, où l'augmentation est en vigueur. Voilà qui pénalise les établissements privés, car le soutien habituel entre les structures hospitalières en cas d'absence de personnel ne pourra plus être assuré si les agents perdent leur prime en venant prêter main-forte dans les structures médico-sociales privées.

je souhaite évoquer les oubliés du Ségur, ces professionnels qui exercent dans les structures accompagnant les personnes handicapées. Les dispositions prévues pour 2022 ne les satisfont pas, car seules certaines professions, qui plus est uniquement sous compétence de l'assurance maladie, verront leur situation évoluer. Aussi, ces structures hospitalières privées comptent sur les orientations issues de la mission Laforcade et souhaitent que l'extension prévue se poursuive, pour permettre de travailler sur l'évolution de la rémunération des autres métiers et des établissements sociaux non concernés par ce protocole. est la suivante : face à l'inquiétude grandissante pour la survie de ces établissements de santé, quelle aide peuvent-ils espérer afin de pouvoir continuer à exister ?

vous évoquez les revalorisations dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les établissements de santé privés. Dès la conclusion des accords du Ségur au mois de juillet 2020, la transposition a été prévue pour les personnels non médicaux, et elle a été mise en oeuvre pour plus d'un million de professionnels. Le complément de traitement indiciaire a été transposé pour les établissements de santé privés, et il en est de même de la revalorisation des grilles de soignants. Si le Ségur de la santé ne prévoyait qu'une revalorisation des médecins de l'hôpital public, le Premier ministre a annoncé au mois de mars dernier une revalorisation salariale des médecins des hôpitaux privés non lucratifs.

personnels soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux qui exercent aujourd'hui dans ces structures percevront une rémunération supplémentaire de 183 euros à compter du 1 janvier 2022. L'impact financier important induit par ces revalorisations sera entièrement pris en compte par l'assurance maladie. Au-delà, monsieur le sénateur, le ministre des solidarités et de la santé, auquel je me joins, souhaitait préciser que les salariés et les agents des établissements médico-sociaux bénéficieront des revalorisations consécutives à la refonte des grilles de rémunérations des personnels paramédicaux- infirmiers, aides-soignants, filières de rééducation

confiés à Michel Laforcade, un premier accord a été signé le 11 février dernier pour revaloriser l'ensemble des personnels non médicaux rattachés aux établissements publics de santé relevant de la fonction publique hospitalière, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur. À la demande du Gouvernement, Michel Laforcade a ensuite poursuivi les discussions avec les organisations syndicales sont intégrés, notamment, les auxiliaires de soins relevant de la fonction publique territoriale. Ces travaux ont abouti à un nouveau protocole signé le 28 mai dernier, qui étend le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l'ensemble des personnels soignants et accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires et contractuels de ces structures financées. Les auxiliaires de soins relevant de la fonction publique territoriale sont donc bien intégrés dans cette mesure et bénéficieront pleinement de cette revalorisation à compter du 1 octobre 2021. S'agissant du secteur privé, le second accord de méthode, signé le même jour, étendra le bénéfice de la mesure socle aux mêmes professionnels et établissements à compter du 1 janvier 2022. Cette revalorisation était indispensable. Le Gouvernement a conscience des attentes légitimes qu'elle a pu créer chez d'autres catégories de personnel. Dans les autres secteurs, toute éventuelle revalorisation doit faire l'objet d'une discussion approfondie avec les conseils départementaux dont dépendent ces politiques. Le Gouvernement reste bien sûr mobilisé et travaille sur ces enjeux. La parole est

Depuis 2019 et, plus récemment encore, depuis la crise sanitaire, les violences conjugales et les féminicides se multiplient : on en dénombre 7 dans le Nord en 2020 et déjà 86 à l'échelon national pour l'année en cours. À la suite du Grenelle des violences conjugales, le bracelet anti-rapprochement permettant l'éloignement des conjoints et ex-conjoints violents devait être généralisé à tous les tribunaux. La France en possède 1 000, mais une poignée seulement est ordonnée par la justice à destination des conjoints violents. Dans les affaires de Mérignac et d'Hayange, les hommes condamnés

selon les chiffres, dans le Nord, seuls 32 bracelets anti-rapprochement ont été déployés, principalement à Douai. Par ailleurs, au mois de juin dernier, les procureurs ont demandé des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales, notamment la création d'assistants spécialisés ou de juristes dédiés à cette cause. Ces postes seraient nécessaires par exemple pour vérifier qu'une mesure d'interdiction d'entrer en contact est bien respectée ou pour prescrire un bracelet anti-rapprochement, si tel n'est pas encore le cas.

Certes, 414 bracelets anti-rapprochement en moins d'un an en France, ce n'est pas encore suffisant, mais cela reste un encouragement fort. Depuis le début du déploiement de la mesure, on dénombre 426 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure au déclenchement d'une alarme, qui ont permis d'éviter des crimes. Il faut rappeler que ce dispositif est déployé de manière opérationnelle dans toutes les juridictions, mais que son attribution dépend des décisions de l'autorité judiciaire.

sont déployés, dont 1 768 sont actifs, et nous venons de décider de porter leur nombre à 3 000, soit une augmentation de plus de 60 % en un an. C'est un instrument de protection efficace. En 2020, il y a eu

3 254 ordonnances de protection ont été délivrées, contre 1 388 en 2017. Comme la question des moyens est également essentielle, le garde des sceaux a décidé de prévoir des emplois supplémentaires spécifiques pour traiter

avoir des informations sur ce qui se passe précisément dans le département du Nord, où la situation est alarmante. Les moyens n'y sont pas à la hauteur de la situation, qui est gravissime.

l'attention du garde des sceaux sur ce qu'on peut appeler un loupé dans la mise en oeuvre de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application concernant les associations d'aide aux victimes. Le décret d'application de la loi de 2019 prévoit

conséquence, des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), qui sont indispensables et expérimentés dans l'accompagnement des victimes de violences, se voient refuser l'agrément

D'importantes subventions sont chaque année allouées à ces structures par le ministère de la justice. Il est exact que, au regard des critères actuellement en vigueur, les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes ne peuvent pas obtenir l'agrément du ministère de la justice, le texte prévoyant que, pour être agréée, l'association doit être en mesure de proposer à toute personne victime d'une infraction pénale

actuellement confiées, autorisera les parquets à saisir les associations spécialisées en matière de violences faites aux femmes pour réaliser des évaluations personnalisées des victimes et pallier ainsi les difficultés que vous avez clairement décrites. La parole

se voir de nouveau attribuer l'agrément pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales et intraconjugales. Je vous remercie de bien vouloir dire de ma part au garde des sceaux que c'est une bonne idée.

Mais force est de constater qu'un certain nombre de services d'accompagnement ne pourront pas survivre aux tensions et aux crises qu'ils connaissent actuellement. Je rappelle enfin qu'une journée d'hospitalisation coûte en moyenne plus de 1 200 euros, une journée de prise en charge à domicile. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour accompagner ces établissements et répondre à la demande croissante des Français de services d'accompagnement à domicile ? La parole est

Nous aurons de plus en plus besoin de ces métiers : des emplois devront être créés par dizaines de milliers pour accompagner nos concitoyens, qui souhaitent massivement vieillir à domicile. Il fallait donc apporter une première réponse aux salariés de la branche de l'aide à domicile : ils l'attendaient depuis quinze

Le coût de cette revalorisation pour les départements, dont relève cette compétence, sera allégé de moitié, et même de 70 % en 2021. C'est historique, tant par les montants mobilisés que par la démarche partenariale engagée. Nous avons besoin d'accompagner toutes les structures du secteur de l'aide à domicile, y compris celles du secteur privé commercial, afin de leur permettre de mieux rémunérer et de mieux former leurs salariés. Il s'agit ainsi de rendre ces emplois d'avenir plus attractifs. C'est pourquoi, comme le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques jours, il sera proposé au législateur de créer un tarif plancher

chargée de l'industrie. Monsieur le ministre, s'il existe une pratique commerciale que nos concitoyens ne supportent plus, c'est bien le démarchage téléphonique non sollicité. Dans mon département, l'Essonne, ils sont nombreux à me demander d'agir pour mettre fin à ce qui s'apparente souvent à du harcèlement. Le nombre d'appels reçus quotidiennement est tel qu'on ne fait plus la différence entre le sondeur qui étudie l'opinion, l'opérateur téléphonique qui tente de récupérer un nouveau client mobile, l'entrepreneur qui propose ses produits, pas toujours innovants, ou encore le cabinet de conseil en investissements immobiliers. À ces pratiques, parfois à la limite de la légalité, s'ajoutent le démarchage par automate d'appel et la fraude aux numéros surtaxés. Cette dernière n'a pas disparu, tant s'en faut, et continue à déstabiliser les publics vulnérables, comme les personnes âgées ou handicapées, ainsi Certes, le législateur est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années pour tenter de juguler ces pratiques, mais force est de constater que la réponse des pouvoirs publics est bien trop faible. Bloctel d'opposition au démarchage téléphonique ne garantit pas de ne pas être contacté et la fraude aux numéros surtaxés continue allègrement à prospérer. En voulant préserver coûte que coûte l'activité des professionnels vertueux, on laisse se développer à la marge des comportements frauduleux qui pénalisent irrémédiablement le consommateur. consommateur. La loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux tarde à produire ses premiers effets. Et pour cause, plusieurs mesures réglementaires prévues par cette loi n'ont toujours pas été prises par le Gouvernement, le décret déterminant les jours, les horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale peut avoir lieu, ainsi que le décret précisant le code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels du secteur. Ma question sera très précise, monsieur le ministre : pouvez-vous m'indiquer l'échéancier de mise en oeuvre des mesures réglementaires que doit prendre le Gouvernement ?

Elle introduit également une interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, où les abus étaient particulièrement prononcés ces dernières années. Elle permet aussi de lutter plus efficacement contre les usurpations de numéros de téléphone, qui complexifient les enquêtes des fraudes (DGCCRF). Nous sommes en cours de finalisation des décrets d'application de cette loi, en particulier du décret qui viendra prochainement encadrer les jours et les horaires auxquels le démarchage téléphonique est autorisé, ainsi que la fréquence des appels. Ce décret, vous le savez, a fait l'objet d'une consultation des parties prenantes durant l'été. La DGCCRF poursuit une action répressive résolue pour sanctionner les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations légales. Ainsi, en 2020, 1 503 établissements ont été contrôlés et ont conduit à sanctionner 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d'opposition au démarchage téléphonique, pour un montant total d'amende de 4,3 millions d'euros, soit le double de l'année 2019. Par ailleurs, une modernisation du service Bloctel est en cours avec un nouveau délégataire et l'interface sera bientôt plus intuitive. Enfin, la lutte contre les fraudes aux numéros surtaxés a été renforcée. La dernière enquête de la DGCCRF a permis de constater que, sur dix-neuf entreprises visitées, sept ne respectaient pas un ou plusieurs points de la réglementation applicable. Vous pouvez compter, madame la sénatrice, sur la mobilisation du Gouvernement en la matière.

Bien que cette mesure aille dans le bon sens, car elle encourage nos agriculteurs à se convertir à l'agriculture biologique, certaines de nos communes, les plus petites, ne peuvent l'appliquer, compte tenu du manque à gagner qu'elle Dès lors, le Gouvernement envisage-t-il une compensation pour les communes mettant en place cette exonération, même conditionnée, de taxe sur le foncier non bâti pour les agriculteurs en conversion biologique, soit de la part d'État, soit de la part de la région ?

initiale de 2009 a permis aux collectivités territoriales d'instaurer, sur délibération, une exonération de taxe foncière au profit des agriculteurs en conversion biologique. Elle visait ainsi à mettre à disposition des collectivités un outil incitatif au développement des surfaces exploitées selon un mode de production biologique. Cette exonération de taxe foncière, prévue à l'article 1395 G du code général des impôts, relève de la seule décision des communes et des Toute compensation de l'État a donc été écartée. L'exposé des motifs de l'article 52 du projet de loi de 2009 le précisait. Le dispositif respectait les principes défendus alors par la commission des finances du Sénat, en vertu desquels les décisions d'allégement d'impôts locaux devaient devaient être prises par les collectivités concernées afin de leur permettre de conserver la maîtrise de l'assiette de leur fiscalité. Par ailleurs, le rapporteur général de ladite commission précisait que les collectivités devaient supporter le coût des allégements afin de préserver leur pleine responsabilité décisionnelle. D'une manière plus générale, il convient de rappeler que, en matière de compensation des pertes de recettes induites par les exonérations ou abattements de fiscalité locale, l'État n'est soumis à aucune obligation de nature juridique. En pratique, lorsque ces exonérations ou abattements résultent d'une décision de l'État, ce dernier fait le choix de compenser les collectivités à l'euro près. Depuis 2017, le Gouvernement l'a fait à la suite de la réforme de la suppression de la taxe d'habitation ou, plus récemment, de celle des impôts de production. À l'inverse, lorsque ces exonérations ou abattements résultent d'une délibération des collectivités, ils ne sont pas compensés par l'État, mais sont à la charge des collectivités elles-mêmes. Conformément à cette pratique, il n'est pas envisagé de revenir sur l'absence de compensation de l'exonération prévue à l'article 1395 G du code général des impôts. Le recours à cette exonération est le fruit d'une décision des collectivités concernées.

une baisse des taux de subvention de cet outil pourtant indispensable à l'aménagement du territoire et à l'équité territoriale. J'ai été alerté par le syndicat mixte Territoire d'énergie Mayenne. Cette autorité organisatrice de la distribution d'électricité d'électricité craint une réduction du volume total des aides alors que le niveau de péréquation prévu pour l'électrification rurale est fortement rationné. Son inquiétude est d'autant plus forte que la Mayenne est un département à dominante rurale, qui compte 27 communes de plus de 2 000 habitants, dont le territoire est couvert à 80 % de terres agricoles- un peu moins de 8 % de la surface est urbanisée -et où la densité de la population est deux fois plus faible que la densité nationale. En laissant 20 % à la charge des collectivités, maîtres d'ouvrage sur les travaux d'électrification rurale, il est garanti, par la péréquation financière, une égalité dans les coûts d'accès au réseau de distribution d'électricité entre les consommateurs ruraux et les consommateurs urbains. La remise en question à la baisse de la participation de l'État est aggravée par la proposition d'établir un lien entre le compte d'affectation spéciale « FACÉ » et le Fonds de péréquation de l'électricité (FPE), qui assure la péréquation des ressources tarifaires au profit de certaines entreprises locales de distribution d'électricité, ce qui accroît les inquiétudes des élus. Les orientations à la baisse de ces taux d'intervention suscitent l'incompréhension des élus de nos collectivités rurales, qui vont voir le niveau de la péréquation financière dont elles bénéficient en matière électrique diminuer, alors qu'il leur est demandé un effort fiscal bien supérieur à celui que doivent dégager les collectivités urbaines dans ce domaine. J'ajoute que les territoires ruraux se voient jouer un rôle décisif dans la transition énergétique. Ma question est simple, allez-vous reconsidérer ce projet de réforme afin de maintenir le modèle de solidarité entre urbains et ruraux et d'assurer un indispensable service de l'électricité de qualité sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones les plus fragiles ? est à M. le ministre délégué. Monsieur le sénateur Chevrollier, Mme la ministre de la transition écologique ne pouvant être présente, elle m'a chargé de vous répondre. Avec le compte d'affectation spéciale « FACÉ » que vous avez décrit, l'État finance des opérations visant à améliorer la qualité de la distribution d'électricité dans les zones rurales et à contribuer à leur transition énergétique. Ces opérations sont sous maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE). Le décret du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale prévoit que le taux de subvention pour chaque aide est fixé par arrêté de la ministre chargée de l'énergie, dans la limite de 80 % du coût du projet. L'arrêté pris le 13 avril 2021 fixe d'ailleurs pour 2021 les taux de subvention à ce plafond. Un travail technique a été engagé avec les représentants de l'administration et des AODE pour évaluer les taux nécessaires à la bonne réalisation des opérations sur chacun des sous-programmes du FACÉ. En fonction des résultats de ce travail, les taux de subvention pour 2022 ou les années ultérieures pourraient évoluer. Il ne s'agit cependant, à ce stade, que d'un examen, afin de s'assurer de la pertinence des taux. Aucune décision sur une éventuelle baisse des taux pour certains types d'opérations n'a été prise. n'a été prise. L'administration sera particulièrement attentive à la bonne prise en compte des surcoûts liés à la ruralité. L'amendement visant à modifier les règles de calcul du Fonds de péréquation de l'électricité qui a été déposé par le Gouvernement lors de l'examen par le Sénat du projet de loi locale a été déclaré irrecevable avant son examen. Le Gouvernement a entendu les inquiétudes des AODE et n'envisage plus de créer de lien entre le FPE et le FACÉ. Le Gouvernement réaffirme son attachement au dispositif des aides à l'électrification rurale, outil crucial pour assurer une bonne qualité de distribution d'électricité sur tout le territoire. Cet attachement se manifeste notamment par le maintien, depuis plusieurs années, d'une aide d'un montant de 360 millions d'euros par an. La parole

du S-métolachlore est un herbicide utilisé pour le désherbage de nombreuses cultures de printemps, notamment le maïs et le soja. Depuis le 1 janvier 2021, ce métabolite fait partie des molécules recherchées dans l'eau mise dans l'eau mise en distribution. L'eau est considérée comme étant non conforme dès que la limite de qualité réglementaire de 0,1 microgramme par litre est dépassée,

trouver des solutions et mettre en place des mesures préventives et curatives. La maîtrise de l'aire de captage d'eau potable est un enjeu. D'ailleurs, l'un des principaux fabricants de produits sanitaires indique que ces produits ne doivent pas être utilisés

des dérogations accordées aux collectivités, notamment celles dont le dépassement est faible ? Enfin, quels accompagnements financiers des collectivités et des agriculteurs envisagez-vous afin de rendre soutenables ces adaptations ?

Vous avez raison, les ressources en eau des captages sont trop souvent contaminées par les pollutions diffuses. La dernière alerte concerne la présence du métabolite du S-métolachlore, herbicide fréquemment utilisé, notamment sur le maïs.

Fermer les captages contaminés ou traiter l'eau ne constituent pas des solutions durables et ont un coût trop important. Restaurer la qualité des eaux à la source doit être la priorité pour assurer l'accès à une eau potable de qualité, à un prix abordable dans la durée. Il existe d'autres solutions efficaces que l'utilisation de ce pesticide, comme le désherbage mécanique. Les financements de la politique agricole commune seront mobilisés pour déployer ces solutions en priorité sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable. Les ministres de l'écologie, de la santé et de l'agriculture ont d'ores et déjà engagé plusieurs actions.

Ils ont également mobilisé l'Anses au mois de mai, en tant qu'autorité de gestion des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et responsable de la phytopharmacovigilance. Il est par ailleurs indispensable que les préfets se saisissent de ce problème et accompagnent plus activement les collectivités. Le Gouvernement va donc leur adresser une instruction afin qu'ils accélèrent la transition agroenvironnementale sur les aires de captage et qu'ils mobilisent l'ensemble des outils disponibles pour reconquérir la qualité de l'eau et prévenir sa dégradation. Ainsi, les collectivités

remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Il est indispensable de laisser du temps à l'ensemble des acteurs de mettre en place ces mesures préventives, voire curatives, et surtout de les accompagner financièrement.

Aujourd'hui, l'exaspération est à son comble. Les riverains sont épuisés par cet enfer routier permanent : le bruit des camions qui montent le col du Bonhomme, la vitesse de ceux qui descendent, les vibrations sur les maisons, l'état de la route et des réseaux souterrains, tout n'est que pollution, contrainte, danger et stress. Ce secteur magnifique est pris en otage par le transit routier. Les conséquences sur l'économie locale et sur l'immobilier sont désolantes. Les longs courriers et les longs discours n'ont rien changé et les riverains se sentent abandonnés. Aujourd'hui, ils expriment une colère légitime et les élus sont démunis. Cela ne peut plus durer. À l'heure où nos concitoyens repensent leurs déplacements, la traversée du Bonhomme devient un enjeu majeur de la politique de transport local. Il faut maintenant trouver des solutions adaptées et pérennes, car notre territoire ne peut plus plus attendre ni se contenter des mesures qui ne règlent pas le problème. Plusieurs comités de pilotage ont été mis en place, sans succès à ce jour. Aujourd'hui, il faut agir rapidement. Ma question est la suivante

La situation évoluera avec l'ouverture de la déviation de Châtenois, opération largement financée par l'État, dont les travaux doivent s'achever en 2023. Cela rendra cet itinéraire plus attractif et soulagera les autres franchissements vosgiens, dont le col du Bonhomme. Dans cette attente, l'État ne souhaite pas voir les poids lourds circuler davantage dans la commune de Châtenois, où les bouchons, vous l'avez dit, sont déjà importants. Brider le trafic local ne semble pas non plus adapté de part et d'autre de la route des crêtes. Cela entraverait l'activité économique des Vosges, alors que les besoins sont réels, notamment pour le transport de grumes. J'ai donc demandé, en cette rentrée, aux services de mon ministère de relancer les travaux du comité de pilotage en lien avec toutes les parties prenantes, dont les collectivités locales et les acteurs économiques. Nous avons, grâce à ces échanges, réussi par le passé à trouver des solutions concrètes, comme la diminution drastique du péage du tunnel Maurice-Lemaire ou la déviation de Châtenois. Je souhaite que ce travail soit poursuivi pour anticiper les futures modalités de franchissement vosgien par les poids lourds au travers de mesures très concrètes.

des transports. Monsieur le ministre, du fait de la crise du covid, la fréquentation ferroviaire s'est effondrée. SNCF Voyageurs a perdu 97 % de son chiffre d'affaires sur le TGV au plus fort de la pandémie. À l'heure de la reprise, la densité des flux de mobilité de la SNCF est centrale, parce qu'il lui faut, stratégiquement et économiquement, accueillir davantage d'usagers et parce que la transition énergétique et environnementale l'impose. Mais patatras ! Le train-train qui lui sied n'est pas au rendez-vous

Avant la crise, la qualité de service de cette ligne était remarquable, mais, aujourd'hui, le niveau de l'offre est dégradé. La forte fréquentation de cette rentrée n'a pas été accompagnée par la réouverture des sillons annulés avant l'été. Il manque la bagatelle de cinq allers-retours quotidiens pour revenir au cadencement de 2019 toutes les trente minutes. Comment expliquer cela ? Comment expliquer à des milliers d'Aquitains que la suppression brutale et incompréhensible de la liaison aérienne Bordeaux-Orly n'ait pas été suivie de l'accroissement mécanique du report modal sur le train ? Que dire des propos sur le nombre de dessertes quotidiennes promis aux collectivités, celles qui ont mis la main au portefeuille pour financer cette ligne voilà quelques années ? SNCF Voyageurs ne se sent plus lié par l'engagement pris lors des négociations originelles avec SNCF Réseau. L'État n'a pas tenu sa parole à cet telle situation n'est pas tenable. Elle est même injustifiable. Monsieur le ministre, comment comptez-vous peser pour inverser la trajectoire et permettre aux usagers de retrouver un niveau de service en rapport avec le prix souvent très élevé du billet qu'ils ont acheté

aux restrictions de déplacement mises en place et au protocole sanitaire. À cet égard, je tiens à saluer l'engagement de la SNCF et de tous ses salariés, qui ont été à pied d'oeuvre chaque jour. Avec souplesse, la SNCF a adapté en permanence le niveau d'offre à la réalité des besoins de déplacements de nos concitoyens. Toutes les adaptations réalisées ont été temporaires. je suis en permanence attentif à ce que le niveau de service ferroviaire soit adapté aux besoins de nos concitoyens. Dès la fin du dernier confinement, l'offre sur l'axe Atlantique Sud-Ouest a été augmentée de 50 % pour faire face à la reprise progressive des voyages. Pendant l'été 2021, l'offre à grande vitesse est remontée à 95 % du niveau de 2019, soit plus de 40 000 places offertes chaque jour. Pour 2022, je peux vous confirmer que le niveau d'offre prévu sur la liaison Paris-Bordeaux s'élèvera à dix-neuf allers-retours quotidiens. Il ne présente donc pas de diminution. Par ailleurs, pour tenir compte des évolutions sur la liaison aérienne Orly-Bordeaux, j'ai missionné Mme la préfète de région, qui a déjà commencé à réunir les acteurs locaux, pour voir si des améliorations routières ou de transports en commun étaient nécessaires, notamment pour faciliter l'accès à la gare bordelaise. Elle me rendra compte dans les prochains jours.

Si l'effet du raccordement au poste source est intégré à l'évaluation environnementale, l'étude sur ce point est souvent insuffisante. Un projet peut être autorisé sans que le tracé du raccordement soit connu. Or il n'est pas sans conséquence pour les territoires traversés.

L'inquiétude est là. Comment peut-on ainsi enterrer des câbles de 20 000 volts sans aucune évaluation préalable des risques sur la santé des personnes et des animaux ? Les élus locaux et les habitants ne sont ni consultés ni suffisamment informés en amont de l'existence et du tracé du raccordement. Pis encore, il n'est souvent pas tenu compte des avis formulés par les élus ni, plus généralement, de l'intérêt des communes traversées. Dans mon département, la Vienne, plusieurs communes n'ont pas eu d'autre choix que d'interdire l'enfouissement de câbles sur leur territoire. On parle beaucoup de décentralisation et d'acceptabilité des projets. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour tenir compte de l'avis des communes concernées ? La parole est à M. Monsieur le sénateur, vous interrogez Mme la ministre de la cohésion des territoires et Mme la ministre de la transition écologique sur les conditions de raccordement électrique des parcs éoliens. Il est important de le rappeler, le développement des énergies renouvelables, dont l'énergie éolienne, est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Les conditions de raccordement électrique des parcs éoliens sont très encadrées. Depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la réglementation exigeante des des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et à une procédure d'autorisation permettant de s'assurer que les risques et inconvénients pour les riverains et l'environnement peuvent être efficacement prévenus. Leur raccordement fait l'objet d'une consultation des maires et des services. Les modalités sont adaptées selon

En application du code de l'environnement, ces schémas sont soumis à évaluation environnementale et font l'objet d'une consultation du public. Pour l'éolien en mer, les possibilités de raccordement sont présentées en même temps que le projet de parc lors de la procédure de participation du public, qui a lieu très en amont de la réalisation du projet. Le raccordement fait de plus l'objet d'une autorisation environnementale, qui donne lieu à une enquête publique et permet aux élus de s'exprimer une nouvelle fois. Il faut le noter, l'arrêté du 17 mai 2001 précise les contraintes techniques qui s'imposent aux gestionnaires de réseau pour tenir compte des risques sur la santé des personnes et des animaux. Enfin, l'occupation du domaine public communal, notamment de la voirie, par les ouvrages électriques fait l'objet de redevances, dont la fixation relève, dans la majorité des cas, de la compétence du conseil municipal. Mes chers

de Dabo une discrimination flagrante en matière d'héritage entre les hommes et les femmes. Cette discrimination provient d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, confirmé par la cour d'appel de Leipzig à l'époque de l'Alsace-Lorraine. Je vous avais interrogée une première fois le 19 novembre en vous demandant pourquoi vous tolériez que certains droits ne puissent pas être hérités par les femmes. Vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai de nouveau posé une question écrite le 5 août 2021. Vous ne m'avez toujours pas répondu. C'est ce qui m'a amené à poser la question orale orale publiée au du 30 septembre 2021. Il vous suffit de lire les questions concernées pour comprendre le problème. Maintenant, j'attends une réponse ! La parole Monsieur le sénateur, ma collaboratrice parlementaire a reçu une demande de prise de contact par mail, sans autre indication- c'était simplement une prise de contact -, le 26 août dernier. le 26 août dernier. À son retour de congé, le 2 septembre, elle a immédiatement répondu à votre message. Vous ne lui avez pas indiqué en retour ce que vous attendiez. Si je comprends bien, vous vous plaignez de ne pas avoir eu de réponse de la part de mon cabinet alors que vous avez adressé des questions au ministère de l'agriculture. Vous savez que je suis ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je ne pouvais donc pas répondre à un message envoyé à un ministère autre que le mien. Sur le fond, vous attirez mon attention sur le régime dit du « bois bourgeois », qui est en vigueur dans les communes de l'ancien comté de Dabo. Les droits d'usage forestier sont un héritage du droit féodal, que le code forestier de 1827 fait perdurer jusqu'à nos jours, nouvelle possibilité de reconnaître de nouveaux droits d'usage dans les bois et forêts de l'État, sous quelque prétexte que ce soit. Parmi ces droits d'usage, il existe un droit dit du « bois bourgeois qui consiste en la délivrance de tronçons d'arbres résineux, et ce par tirage au sort annuel, au bénéfice des usagers remplissant les conditions de délivrance. Datant de l'Ancien Régime, ce droit ne reconnaît la qualité d'usagers qu'aux hommes. Malheureusement, ce n'est pas le seul. Il est effectivement très étonnant que, de nos jours, persiste un dispositif excluant les personnes de sexe féminin non mariées. Seules les veuves peuvent conserver le droit acquis par leur mari, dans une mesure réduite, jusqu'à leur remariage. De telles dispositions portent clairement atteinte au principe de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Vous pouvez donc imaginer combien j'aurais été heureuse de répondre à votre question.

je trouve tout de même stupéfiant que la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit pas choquée par une

de l'agriculture et de l'alimentation. Pierre angulaire de la future politique agricole commune (PAC), le ou Pacte vert suscite de vives inquiétudes chez nos agriculteurs. En renonçant à l'horizon 2030 à 10 % de la surface agricole utile européenne, tout en diminuant de 50 % les pesticides et en quadruplant les terres bio, la nouvelle PAC pénalisera immanquablement l'agriculture traditionnelle, qui représente pourtant l'essentiel de la production européenne.

! Ce se traduira aussi par une baisse sans précédent de la production agricole européenne : de 12 % d'ici à 2030 selon le ministère américain de l'agriculture de 5 % à 15 % selon l'étude d'impact des stratégies « De la ferme à la fourchette » et « Biodiversité », rendue publique discrètement en plein coeur de l'été par la Commission européenne, après plus d'un an de tergiversations. Le annonce donc la décroissance et la fin de la souveraineté alimentaire de notre continent. Comment la France entend-elle empêcher un tel désastre et sauver notre modèle agricole traditionnel ? La parole est à

comporte un programme de travail en termes de stratégies et de propositions législatives. Il propose des objectifs chiffrés à l'horizon 2030 en termes de part de la surface consacrée à l'agriculture biologique, soit 25 % à l'horizon 2030, ou de réduction de l'usage et des expositions aux produits phytopharmaceutiques, soit une baisse 50 % à l'horizon 2030. Une étude d'impact partielle a enfin été publiée au coeur de l'été par la Commission. Son bilan montre que, sans action forte en politique commerciale, l'on risque une décroissance verte. Or ce n'est l'intérêt de personne. Je regrette le manque de transparence de cette publication tardive de l'étude, après l'accord sur la réforme de la PAC. Les propositions législatives annoncées dans les stratégies doivent être présentées par la Commission dans l'année à venir.

de manière adaptée et que toutes les politiques européennes y contribuent. Il s'est aussi battu pour une articulation avec les objectifs du Pacte vert, mais dans le respect des objectifs propres que le traité fixe à la PAC : assurer notre souveraineté alimentaire

Monsieur le ministre, la forêt a un rôle central dans la construction de l'identité de notre pays. Elle participe à la fois à son histoire, à son actualité et à son avenir. Il s'agit d'un patrimoine naturel aux enjeux économiques, culturels et de loisirs. Sur le plan environnemental, la forêt demeure le plus riche des réservoirs de biodiversité et permet chaque année l'absorption de 15 % des émissions françaises de carbone. Aujourd'hui, la filière forêt-bois est en crise pour plusieurs raisons, liées notamment au changement climatique et aux invasions de parasites, mais surtout à l'obsession de la rentabilité rapide, qui a abouti à des exportations massives des grumes françaises vers l'Asie et les États-Unis. La crise sanitaire et la reprise économique bien commun est reconnu de longue date par le vicomte de Martignac. En effet, dans son exposé des motifs du projet de code forestier de 1826, celui-ci considérait déjà : « La conservation des forêts est l'un des premiers intérêts des sociétés et, par conséquent, l'un des premiers devoirs des gouvernements. » Ainsi, la gestion de forêts ne peut reposer que sur des logiques de long terme, dans lesquelles les communes forestières jouent un rôle reconnu. Or le Gouvernement envisagerait une nouvelle contribution des collectivités au financement de l'Office national des forêts (ONF), laquelle aurait des conséquences sur les budgets des communes, qui seraient une fois encore fragilisées. Ce n'est pas acceptable dans le contexte actuel, alors que les communes ont déjà contribué au soutien de l'ONF. De même, il est dangereux de démanteler le service public forestier en le dépouillant de ses agents et de moyens. La forêt exige une gestion planifiée et adaptée à la spécificité de chaque milieu. L'expertise acquise par les agents de l'ONF depuis plus de cinquante ans et leur rôle de conseil auprès des décideurs locaux sont indispensables et ne sauraient être sacrifiés. Aussi, je vous demande de bien vouloir envisager de revenir sur ce projet d'augmentation des contributions des communes forestières tout en maintenant les moyens de l'ONF pour la gestion de nos forêts. La parole Monsieur le sénateur, le Gouvernement est attaché à la pérennité de l'ONF et entend conserver l'unité de gestion des forêts publiques domaniales et communales par l'Office. Pour mener une politique forestière ambitieuse et de développement des usages du bois, l'État a besoin d'un ONF fort et performant au regard des défis que rencontre la forêt face au changement climatique et de son potentiel en termes de valorisation du bois et d'atténuation du changement climatique. La gestion durable et multifonctionnelle est au coeur du modèle de l'ONF et doit le rester. Ce principe est un élément central du nouveau contrat entre l'État et l'ONF pour la période allant de 2021 Pour autant, l'ONF connaît depuis plusieurs années une situation financière déséquilibrée, ce qui appelle des réponses conjoncturelles, mais aussi structurelles, notamment sur son modèle de financement. Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de renouveler, dans le cadre du contrat État-ONF pour les années 2021 à 2025, sa confiance en l'Office, tout en engageant des mesures importantes visant à lui redonner des perspectives soutenables. L'État maintient le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'ONF et réaffirme qu'il n'existe aucun projet de privatisation. Ce contrat conforte les missions d'intérêt général portées par l'ONF et consacre la notion de prise en charge à coût complet de ses missions, quel qu'en soit le commanditaire. L'État revalorise substantiellement ses missions à hauteur de plus de 12 millions d'euros dès cette année 2021 et de 22 millions d'euros en 2024, ce qui portera le financement par l'État de ses missions à 55 millions d'euros par an. En outre, le Gouvernement décide de mobiliser 60 millions d'euros complémentaires dès cette année et sur les deux années à venir, à raison de 30 millions d'euros en 2021, de 20 millions d'euros en 2022 de 10 millions d'euros en 2023 pour soutenir l'établissement tout en renforçant la subvention d'équilibre. Cela vient en plus des 140 millions d'euros de versement compensateur annuel. dans le cadre du volet forestier du plan de relance, une dotation de 30 millions d'euros a été allouée pour 2021 à l'ONF afin de financer la reconstitution des forêts domaniales atteintes par les crises sanitaires.

Cette bactérie, présente dans le département de l'Aude, et plus particulièrement concentrée sur le territoire de l'agglomération de Carcassonne, est phytopathogène. Elle est transmise et véhiculée par des insectes vecteurs. Elle possède un large spectre de végétaux hôtes et peut s'attaquer à plus de 300 espèces végétales. Par arrêté préfectoral du 19 février 2021, il a été demandé aux collectivités concernées de réaliser les actions d'assainissement des foyers pour en limiter au maximum la propagation.

Face à l'enjeu sanitaire, économique et social, la mobilisation des collectivités audoises concernées est totale dans la réalisation des interventions. Je tiens ici à les saluer. Mais le financement est problématique, car les moyens n'étaient pas inscrits dans la loi de finances pour 2021. À ce jour, aucun fonds n'est prévu pour aider les collectivités dans la mise en oeuvre des mesures. Le programme d'indemnisation élaboré agricole de mutualisation du risque sanitaire environnemental pour les préjudices relatifs à la destruction de végétaux et aux restrictions de circulation n'est pas ouvert aux collectivités territoriales. Des modalités de soutien financier

La bactérie est présente dans douze communes. Les services de l'État mettent en place des mesures de lutte afin de l'éradiquer, ainsi qu'une surveillance renforcée, conformément au règlement d'exécution du 14 août 2020. Ce règlement, dont la mise en oeuvre est détaillée dans le plan national d'urgence, exige un enlèvement immédiat des végétaux infectés, ainsi que des végétaux sensibles à la bactérie bactérie dans la zone infectée, qui correspond à une zone de cinquante mètres de rayon autour d'un végétal contaminé. L'État a pris en charge la gestion du premier foyer détecté en pépinière en 2020. Un programme d'indemnisation de la section pépinières et horticulture a été depuis déposé, afin d'indemniser l'opérateur professionnel concerné. Les végétaux contaminés trouvés dans les autres zones infectées en 2020 ont été arrachés par les propriétaires et, afin d'accélérer leur destruction, une entreprise est intervenue aux frais de l'État au printemps 2021 pour les végétaux restant à détruire. La destruction des végétaux trouvés contaminés en 2021 est en cours. Les services de l'État sont pleinement mobilisés pour mettre en oeuvre les mesures d'éradication et sensibiliser l'ensemble des propriétaires sur leurs obligations au travers de plusieurs canaux de communication.

pour la réalisation des mesures de destruction chez les particuliers. Cependant, la situation en Occitanie est bien différente de celle que l'on observe en région PACA : de nombreux foyers sont situés en zones semi-naturelles et nécessitent parfois des travaux de grande ampleur. Ainsi, vingt et une zones infectées sur les cinquante-neuf concernent à ce stade des collectivités. Au-delà des mécanismes d'indemnisation possibles et du marché déjà attribué pour la prise en charge des arrachages chez les particuliers, les services du ministère chargé de l'agriculture travaillent à d'autres pistes afin d'accompagner les collectivités.

ASA. Face à l'épidémie, il était indispensable de protéger les agents les plus vulnérables. Mais, aujourd'hui, à l'issue du déconfinement, la question des agents dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail

Les nouvelles dispositions parues récemment prévoient là encore de nombreuses exceptions, laissant penser que le dispositif est amené à perdurer. Par manque de personnel, certaines communes doivent désormais sous-traiter leurs travaux, alors qu'elles prennent en charge le salaire de leurs fonctionnaires, et ce sans compensation de l'État.

quelles modalités ? Les congés non pris durant cette période sont-ils perdus ou reportés ? Enfin, quelles sources de financement les collectivités peuvent-elles mobiliser pour maintenir un équilibre financier ? Pour ne prendre qu'un exemple, madame la ministre, j'évoquerai le cas d'un agent en attente d'une greffe et fort probablement vacciné. Il a été durant de longs mois en ASA et non en arrêt maladie.

Monsieur le sénateur Burgoa, l'amélioration de la situation sanitaire a conduit le Gouvernement à faire évoluer très récemment le dispositif de prise en charge des agents territoriaux considérés comme vulnérables, susceptibles de développer des formes graves d'infection au covid-19. Il convient de distinguer la situation des agents vulnérables sévèrement immunodéprimés de celle des agents vulnérables qui ne le sont pas.

ainsi que lorsqu'ils justifient d'une contre-indication à la vaccination. Cette prise en charge spécifique des agents vulnérables est effectuée à leur demande, sur présentation à l'employeur territorial d'un certificat établi par un médecin. Lorsque l'employeur estime que la demande de placement en autorisation spéciale d'absence n'est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l'agent est affecté n'est pas susceptible d'exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail, qui se prononce sur l'exposition à de fortes densités virales du poste et vérifie la mise en oeuvre des mesures

Enfin, les congés annuels des agents vulnérables placés en ASA sont posés dans les conditions de droit commun. Pour ce qui concerne les congés non pris, l'employeur peut, le cas échéant, reporter la date limite à laquelle ils peuvent être posés. Les agents territoriaux conservent en outre la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps dans les conditions de droit commun.

la fermeture de son usine de reconditionnement de pièces détachées à Choisy-le-Roi, dans l'Est parisien, et son transfert à Flins, dans l'Ouest parisien. Cette cessation d'activité est une perte lourde pour le Val-de-Marne, qui voit ainsi partir un site industriel installé depuis plus de soixante-dix ans, avec les emplois qui lui sont liés. Sans baisser les bras, les acteurs locaux- le maire Tonino Panetta en tête, le département, la région et la chambre de commerce et d'industrie -ont engagé

Les premiers résultats de cette étude seront présentés au début de l'année prochaine, mais les premières analyses montrent tout l'intérêt de cette démarche et de ce projet.

afin d'en faire la première usine dédiée à l'économie circulaire de la mobilité. Dans le cadre de ce projet, Renault a décidé de rapatrier à Flins les activités jusqu'ici réalisées à Choisy et de procéder à la fermeture du site. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan de réduction des coûts et de la stratégie révisée de Renault, a fait l'objet d'une attention particulière de l'État, actionnaire de l'entreprise, plus précisément concernant l'avenir des salariés et l'enjeu de préservation de l'activité en France. Renault a signé le 25 mai 2020 un accord avec les organisations syndicales qui encadre les modalités de transfert de l'activité et le reclassement de la totalité des personnels selon trois options options : le transfert vers Flins, le reclassement interne au sein du groupe ou le départ de l'entreprise avec un accompagnement pour reclassement. La majorité des salariés a choisi de poursuivre au sein du groupe, à Flins. Cela témoigne de la pertinence du projet et de l'intérêt d'une activité qui pourra garantir la pérennité de l'emploi. Enfin, Renault s'est engagé, une fois la situation des salariés réglée, à travailler avec les élus locaux

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Cardon, vous le savez, l'accompagnement des jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance fait partie des priorités du Gouvernement. Il mobilise depuis maintenant plusieurs années l'attention du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et d'un grand nombre d'acteurs publics, associatifs ou privés. Cette question est centrale depuis la présentation de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, qui a conduit au déploiement d'actions nationales en faveur de l'insertion professionnelle et de l'autonomie. J'en rappelle quelques-unes : automatisation des bourses de l'enseignement supérieur à l'échelon le plus élevé, soit 680 euros par mois, et accès prioritaire au logement étudiant signature en novembre 2020 d'un accord-cadre avec l'Union nationale des missions locales, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes et la Convention nationale des associations de protection de l'enfant pour mobiliser tous les acteurs les acteurs en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes, un accompagnement personnalisé dès l'âge de 17 ans ; accès automatique, depuis janvier 2021, à la garantie jeunes pour un accompagnement professionnel renforcé et à une aide financière de 500 euros par mois-

qu'il bénéficiera d'une solution pérenne et adaptée. C'est ce qui a conduit l'Assemblée nationale, dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, au vote de l'amendement que vous avez mentionné. En l'occurrence, la question du lien entre les conseils départementaux et les missions locales avait été travaillée bien en amont de ce vote, ce vote, comme en attestent les initiatives que je viens de rappeler. L'accord de 2020, en particulier, construit à partir de bonnes pratiques existantes localement, avait permis de faciliter, d'améliorer et de pérenniser la coordination entre les acteurs de l'aide sociale et de l'insertion. Dans chaque territoire, il permet depuis de promouvoir et d'assurer l'accompagnement des jeunes avant leur majorité, de sécuriser les parcours des jeunes mineurs relevant de la protection de l'enfance jusqu'à leur majorité et de systématiser par des partenariats renforcés l'anticipation des sorties de l'ASE. Il faut conclure ! Vous le voyez donc, toutes ces mesures ont pour objectif d'assurer la protection de ces jeunes. La mise en oeuvre

Depuis la démission du docteur Maurice Raphael en septembre 2020, aucun médecin senior n'a été recruté pour le remplacer au poste de chef de service. À la suite de son départ, onze autres urgentistes ont également quitté l'hôpital et tous les cadres de santé sont partis, tant les conditions de travail y sont déplorables. Le docteur Raphael avait maintes fois alerté sur les dysfonctionnements de ce service. Rien n'a été fait La démission de ce médecin expérimenté, que j'ai rencontré et qui avait véritablement le service public chevillé au coeur, a été le symbole du malaise régnant aux urgences et, plus largement, dans tous les services de cet établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Ce sont des médecins d'autres services qui viendront en aide aux urgences, alors qu'ils ne sont pas urgentistes ! Au regard de cette situation catastrophique, les recrutements se font rares. L'établissement n'est plus assez attractif pour les professionnels. Le service des urgences de l'hôpital Bicêtre est en danger et les patients risquent de l'être aussi. Les professionnels confient eux-mêmes qu'ils n'enverraient pas des proches s'y faire soigner ... Madame la ministre, que compte faire M. Véran face à cette situation catastrophique ? La

Depuis plusieurs années, la situation du service des urgences de l'hôpital Bicêtre appelle notre attention. Une démarche de restructuration profonde a été entamée afin de mettre fin aux difficultés de cette structure. Cette démarche vise à retrouver un fonctionnement optimal et une qualité de vie au travail en phase avec l'attractivité et la renommée de l'établissement. L'ARS d'Île-de-France est mobilisée pour accompagner ce changement et apporter son appui à l'AP-HP. En novembre 2019, l'ARS et l'AP-HP ont signé le premier contrat « zéro brancard pour les patients en attente d'hospitalisation » de la région. L'Agence a validé entièrement la feuille de route élaborée par les professionnels de santé des urgences et la communauté médicale de l'hôpital Bicêtre. À cette occasion, une aide de 500 000 euros a été débloquée et 22 lits supplémentaires de gériatrie aiguë ont été créés au sein de l'établissement. Malgré le retrait d'agrément pour l'accueil des internes, le chef de service nommé au printemps dernier a d'ores et déjà pu procéder à des recrutements et à des changements d'encadrement et d'organisation permettant de répondre aux demandes d'amélioration formulées. L'ARS a proposé de mettre en place et de piloter un comité de suivi mensuel, associant les syndicats d'internes, l'AP-HP et les coordonnateurs des filières de médecine générale et d'urgences. Ce comité permettra de suivre l'amélioration des conditions d'accueil, de travail et de formation des internes, l'objectif étant de permettre au service de retrouver son agrément. Pour les internes qui prennent en charge la permanence des soins aux urgences, une liste de critères et une charte de qualité ont été établies et partagées ; un premier point de situation sur les améliorations apportées par l'établissement a été tenu. Comme vous le voyez, nous soutenons fortement l'établissement, en concertation avec l'ensemble des professionnels de santé concernés, pour que le service des urgences retrouve toutes ses capacités et son attractivité.

qui viennent d'apprendre le prochain départ à la retraite de l'un de leurs trois médecins généralistes. Ce médecin a une patientèle de 1 600 personnes environ, pour lesquelles aucune solution ne se dessine, les deux autres médecins, débordés, ne pouvant plus prendre de nouveaux patients. Face à cette situation, le maire est pleinement mobilisé ; il cherche, à ce jour sans succès, à aider à l'installation d'un nouveau médecin et souhaite y participer financièrement. Il a contacté à plusieurs reprises la préfecture de la Loire et l'ARS, qui n'ont pu lui apporter de réponse satisfaisante quant aux moyens à mettre en oeuvre. Surtout, il a appris que le classement par l'ARS en 2018 de sa commune en zone de vigilance ne lui permet pas d'attribuer des aides destinées à favoriser le maintien de professionnels de santé sur son territoire, en application du code de la santé publique. Seules les communes classées en zone d'intervention prioritaire sont concernées. Face à une telle situation de pénurie, ne serait-il pas envisageable de revoir ce classement ?

À cet égard, les consultations avec la conférence régionale de santé et de l'autonomie et la commission spécialisée pour l'organisation des soins se poursuivent. Sans avoir attendu ce nouveau zonage, l'ARS, en lien avec l'assurance maladie, travaille depuis quelque temps à la structuration des soins de premier recours, est indispensable quand on sait que la jeune génération de professionnels de santé- médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou autres -souhaite avant tout bénéficier d'un exercice coordonné et travailler en pluriprofessionnalité. L'ARS accompagne depuis plusieurs années les projets de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et de centres de santé (CDS), afin de diversifier

de la Loire compte aujourd'hui une quarantaine de MSP et de CDS. Une MSP a d'ailleurs été créée en juillet 2018 dans la commune de Saint-Martin-la-Plaine. Par ailleurs, et afin de faciliter l'installation de nouveaux professionnels, l'ARS a oeuvré pour le développement de la maîtrise de stage, afin de faire découvrir le département aux futurs médecins généralistes et leur permettre de nouer les contacts qui faciliteront leur installation. C'est un succès, puisqu'on estime que trois quarts des maîtres de stage ont réussi à trouver des remplaçants réguliers ou occasionnels grâce à ce dispositif. Aujourd'hui, l'ARS, en lien avec l'assurance maladie, poursuit ses travaux de structuration de l'offre de soins de premier recours en accompagnant les professionnels de santé dans le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), lesquelles permettent de créer des passerelles entre la ville et l'hôpital. Deux CPTS ont d'ailleurs vu le jour dans le département de la Loire en 2020. Nous allons enfin accompagner financièrement les primo-installations

en mode « hyper-ambulatoire ». J'ai reçu au printemps dernier des chirurgiens orthopédistes responsables de centres pilotes, qui ont attiré mon attention

Mme la ministre déléguée. Madame la présidente Catherine Deroche, comme vous le relevez dans votre question, les prises en charge chirurgicales impliquent une garantie totale de sécurité et de qualité pour le patient. Les organisations pour la pratique de la chirurgie ambulatoire en France sont variées, les modèles s'adaptant aux spécialités des territoires. Il peut d'abord s'agir d'une unité de chirurgie ambulatoire au sein d'un établissement de santé pratiquant également l'hospitalisation avec nuitées. Cette unité peut être intégrée au site géographique de l'établissement pratiquant l'hospitalisation complète ou être située sur un site géographique différent : on parle alors de centre indépendant de chirurgie ambulatoire. Ce premier modèle est le plus répandu en France. Les établissements de santé ne pratiquant que la chirurgie ambulatoire, ambulatoire, dénommés en pratique « centres autonomes de chirurgie ambulatoire », constituent un autre modèle. Enfin, que vous évoquez est pratiquée par une structure qui ne constitue pas un établissement de santé- il peut s'agir d'un cabinet de ville, par exemple -, mais dont l'environnement chirurgical se rapproche tout de même de l'environnement hospitalier en termes de normes. Ce modèle Ce modèle est très développé aux États-Unis, mais peu en France à ce jour. Ces cabinets doivent obtenir une autorisation de chirurgie ambulatoire et donc disposer d'un secteur opératoire et du personnel adapté. En outre se pose la question de la réalisation de certains actes chirurgicaux en dehors des blocs opératoires, ce qui permet de rationaliser leur utilisation et les ressources humaines. L'évolution des techniques, notamment anesthésiques, peut en effet permettre, pour certains actes, une prise en charge hors bloc, mais dans un environnement à définir. la communauté scientifique est essentiel pour préciser ces évolutions et déterminer si un acte chirurgical peut se pratiquer en dehors d'un bloc opératoire. À ce jour, l'expérimentation fondée paraît constituer le vecteur idéal pour envisager à la fois de nouvelles organisations sur cette thématique et un modèle financier adapté, dans un cadre sécurisé, avec une évaluation externe qui, le cas échéant, permettra d'adapter la réglementation.

En effet, certaines communes particulièrement dynamiques ont vu leur population augmenter de façon très importante depuis 2016. C'est le cas notamment du sud du département du Tarn-et-Garonne, qui profite de sa proximité avec l'agglomération toulousaine. De très nombreuses communes sont concernées. L'exemple de la commune de Pompignan est particulièrement frappant. La population légale au 1 janvier 2017 était de 1 484 habitants. Elle est aujourd'hui estimée par la mairie à plus de 2 000 habitants, soit 25 % de plus, bien loin de l'estimation de la population annuelle faite par l'Insee. Bien évidemment, cette très forte évolution n'a pas été prise en compte dans le calcul de la DGF, alors que la commune de Pompignan a effectué dans le même temps les investissements nécessaires pour l'accueil de cette nouvelle population. La situation devient même ubuesque lorsque l'administration fiscale rappelle à l'ordre la commune pour mauvaise gestion, ses charges ayant bien évidemment augmenté

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Pierre-Antoine Levi, vous le savez, la population constitue le principal critère de répartition des concours financiers de l'État aux collectivités. collectivités. La population prise en compte dans les calculs est issue du recensement effectué par l'Insee. Les procédures de recensement sont fixées par la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. Celle-ci prévoit notamment qu'un décret authentifie chaque année les chiffres des populations recensées. Seules ces données disposent de la fiabilité nécessaire à la répartition des dotations de l'État. Il ne serait en effet pas possible de fonder ces répartitions sur des données estimatives, sauf à risquer de remettre en cause la fiabilité des calculs, ainsi que l'égalité de traitement entre les collectivités. En raison du contexte sanitaire, l'Insee a annoncé le report à 2022 de l'enquête de recensement prévue initialement pour janvier et février 2021,

Les nombreuses conséquences sociales, économiques et financières de cette décision sont encore perceptibles. La fermeture de nos stations a nécessité la mise en place de mesures de soutien inédites. Je ne peux que me réjouir des divers

Si les aides économiques et financières sont essentielles, leurs effets sur l'activité ne doivent pas être enrayés par des mesures sanitaires trop restrictives, tant pour les professionnels que pour les touristes. De plus, la crise sanitaire a créé un véritable déficit de saisonniers, qui met en péril la mise en mouvement de nos stations de sports d'hiver lors de la saison à venir nous manquerons sans doute de main d'oeuvre. Les modalités de réouverture doivent permettre une reprise sereine de l'activité et favoriser l'attractivité des territoires de montagne. Dans ce contexte, quelles mesures sanitaires seront applicables aux stations de sports d'hiver ?

la gestion de services ou d'équipements publics en régie par les collectivités compte parmi les modalités d'aménagement du territoire. Elle permet aux élus locaux d'intervenir là où le fonctionnement spontané de l'économie de marché n'assure pas aux habitants des services complets, accessibles à bas coût et maillant tout le territoire. Le Gouvernement y est donc très attaché et surveille avec attention les effets de la crise. Après la clôture des comptes de 2020, nous avons constaté que les recettes tirées de leur tarification avaient baissé de 17 %, alors que les recettes communales n'ont, dans leur ensemble, diminué que de 1,8 %. Ce phénomène touche un nombre restreint de collectivités, notamment celles qui portent des équipements structurants, tels que des piscines, des thermes

équipements sportifs, régies thermales, parcs de stationnement, salles de spectacles, services scolaires et périscolaires, etc. Le décret d'application doit passer au comité des finances locales le 19 octobre et les paiements seront effectués dans la foulée de sa publication. Par ailleurs, l'État a soutenu les régies gérant des remontées mécaniques, lesquelles ont reçu les mêmes aides que les entreprises privées. Dans les Hautes-Alpes, seize exploitants ont ainsi bénéficié d'aides,

Madame la ministre, il y a un an ou presque débutaient les concertations du Fontenoy du maritime. Menées avec l'ensemble de l'écosystème français, elles ont pour ambition de faire de la France l'une des dix premières nations du mondial d'ici à la fin de la décennie. Lors des Assises de l'économie de la mer, qui se sont tenues les 14 et 15 septembre derniers à Nice, la ministre de la mer, Annick Girardin, les armateurs de France et le Cluster maritime français ont pris un engagement commun. Une série de mesures ont ainsi été annoncées. Elles visent à faciliter le financement et le verdissement de la flotte contrôlée par les compagnies maritimes françaises, à améliorer le parcours et la carrière de nos marins et, plus largement, à soutenir le pavillon français, grâce notamment à la création d'une aide à l'emploi maritime ou à l'organisation d'une réflexion sur le dumping social maritime dans le cadre de la prochaine présidence française du Conseil de l'Union européenne. oeuvre ces engagements et asseoir notre position dans le commerce mondial, la France peut, et doit, s'appuyer sur ses territoires ultramarins. En effet, 97 % de ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive et d'espace maritime sont liés à ces inutile de préciser que les concertations du Fontenoy du maritime et les annonces des Assises de la mer ont été attendues et scrutées avec attention dans les outre-mer. : premièrement, pouvez-vous nous donner le calendrier de mise en oeuvre des mesures qui viennent d'être annoncées ? Pouvez-vous également préciser les propositions sur lesquelles vous travaillez et qui pourraient encore être retenues dans le cadre de ces concertations ? quelles retombées en termes d'emploi, de financement et de formation les territoires d'outre-mer doivent-ils espérer ? La parole

travail de consultation a eu lieu dans le cadre du Fontenoy du maritime, vous l'avez dit. Vous avez également rappelé les annonces faites par le Président de la République lors des Assises de l'économie de la mer à Nice, le 14 septembre dernier. Une spécialité maritime sera créée au sein du service public au sein du service public de l'emploi. D'ici à la fin de l'année, nous définirons une stratégie d'accompagnement des parcours professionnels des marins. Avec plus de trente-huit implantations territoriales, dont une en Guadeloupe,

maritime (ENSM) et nous augmenterons les promotions d'une cinquantaine de marins. Un travail pourra aussi être engagé avec les bassins de recrutement ultramarins. De plus, et c'était attendu, le Président de la République a validé la simplification des critères d'éligibilité au suramortissement vert.

en général. Je pense notamment aux 175 millions d'euros du plan de relance qui seront consacrés au verdissement des grands ports maritimes et des ports autonomes, dont 23,1 millions d'euros sont dédiés aux outre-mer. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, auteur

Les mégalithes sont, après les grottes ornées, les plus anciens monuments historiques de France. Le dolmen de Saint-Paul a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques dès 1889, ce qui montre son intérêt patrimonial patrimonial majeur. Je me réjouis de l'intérêt que vous-même et le maire de Sainte-Cécile-du-Cayrou portez à ce monument. Les dispositions du code du patrimoine fixent le régime juridique applicable au titre des monuments historiques et de l'archéologie.

territorialement compétente. Par ailleurs, les services régionaux de l'archéologie pourront prescrire la réalisation préalable d'une opération archéologique en lien avec le projet de restauration. Le propriétaire n'a en revanche aucune obligation de permettre ou de faciliter l'accès du public au monument.

d'une décision publique ou si cela suppose une décision du particulier. Peut-être peut-on regretter, même si l'on comprend bien qu'il s'agit d'une propriété privée,